La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la désignation des membres de deux missions d'information. En application de l'article 8 du règlement, les listes des candidats remises par les groupes politiques pour la désignation des membres de la mission d'information sur le thème Excellence de la recherche/innovation, pénurie de champions industriels : cherchez l'erreur française » et de la mission d'information sur « L'exploration, la protection et l'exploitation des fonds marins : quelle stratégie pour la France ? » ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du mercredi 19 janvier prochain, après les questions d'actualité au Gouvernement, de la deuxième lecture de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. Acte est donné de cette demande. Nous pourrions prévoir une discussion générale de quarante-cinq minutes. La commission des affaires sociales se réunira pour examiner le rapport et le texte mercredi 12 janvier, au matin.

lois n'a pas adopté le texte de la proposition de loi relative à la commémoration de la répression d'Algériens le 17 octobre 1961 et les jours suivants à Paris,

Dans la discussion générale, la parole est à M. Rachid Temal, auteur de la proposition de loi.

Le Président de la République, le général de Gaulle, a présidé, ce jour, une séance du Commissariat général au plan sur des investissements publics à caractère social, le quatrième Plan devant être soumis au Parlement pour adoption dans un mois. Si les « événements d'Algérie », comme l'on dit alors pudiquement, sont une réalité pour nos compatriotes, avec de la violence et des attentats des deux côtés de la Méditerranée, la France est une démocratie avec des institutions qui fonctionnent.

Ce mardi 17 octobre 1961, à l'heure où des millions de Français se préparent à passer à table, quelques milliers de nos compatriotes, des Français musulmans d'Algérie- c'est le nom officiel depuis la Constitution de 1946 -s'habillent chaudement pour sortir de leur bidonville ou de leur chambre d'hôtel et rejoindre une manifestation pacifique. Cette manifestation est interdite. C'est un fait. Dès lors, personne ne peut contester la présence des forces de police ni même les arrestations. Pour autant, on peut s'interroger sur ce couvre-feu qui concerne uniquement certains de nos compatriotes, en raison de leur statut de « Français musulmans d'Algérie ». Pour eux, le sentiment d'être des Français de seconde zone existe bel et bien. Ce qui

Chacun peut revoir sur les quelques photos existantes les regards des manifestants arrêtés, parfois ensanglantés : ce sont des regards de peur et de douleur. De Brunet à Einaudi, en passant par le rapport Mandelkern, pour ne citer qu'eux, que pouvons-nous dire ? Quelque 20 000 manifestants se retrouvent ce soir-là sur trois zones à Paris, face aux forces de police : le pont de Neuilly, un axe Grands Boulevards-Opéra-place de la République et le boulevard Saint-Germain, à quelques centaines de mètres de notre hémicycle. Plus d'un manifestant sur deux sera arrêté ce soir-là- un taux d'arrestation rare, convenons-en.

le poste central Opéra, le commissariat central du troisième arrondissement et d'autres commissariats à Paris et autour de Paris. Comment expliquer que, parmi ces manifestants et personnes appréhendés, nous puissions compter plusieurs centaines de blessés et plusieurs dizaines de morts ?

La proposition de loi relative à la commémoration de la répression d'Algériens le 17 octobre 1961 et les jours suivants à Paris que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui s'inscrit dans une histoire déjà longue, mais inaboutie. Madame la secrétaire

et reconnaît les responsabilités clairement établies ». Aujourd'hui, il est demandé au Sénat de faire un nouveau pas, d'être une nouvelle fois au rendez-vous de l'histoire. Le travail de mémoire est nécessaire pour rassembler les Français.

à la mémoire des harkis, à la mémoire des appelés du contingent, à la mémoire de l'immigration algérienne : toutes ces mémoires sont complémentaires et nullement concurrentes. Veillons à ne pas les opposer.

la commission des lois n'a pas adopté le texte de la proposition de loi relative à la commémoration de la répression d'Algériens le 17 octobre 1961 et les jours suivants à Paris, et ce pour plusieurs raisons. Je rappelle qu'il s'agit d'un texte symbolique et mémoriel, car les événements de l'époque sont soit couverts par l'amnistie décidée à la fin de la guerre d'Algérie, soit prescrits. La manifestation du 17 octobre 1961 en tant qu'événement singulier, ses causes et ses suites font l'objet d'un important travail historique depuis 1985 et la parution du premier ouvrage sur ce sujet. La recension opérée par deux historiens britanniques ne relève pas moins de deux cents articles consacrés spécifiquement au 17 octobre 1961. Ce travail important rompt avec l'occultation de l'événement, qui, pour des raisons diverses, a touché l'ensemble des acteurs de l'époque. a aussi pu être conduit grâce à l'ouverture des archives de la préfecture de police et de la justice décidée au mois d'octobre 1997 après le procès de Maurice Papon. En effet, sa responsabilité dans la répression de la manifestation en tant que préfet de police de Paris avait été évoquée devant le tribunal. Si les archives n'avaient pas été ouvertes à l'époque, il aurait fallu attendre 2021, soit encore vingt-cinq ans, pour qu'elles deviennent consultables. Parallèlement, un travail mémoriel entrepris par des associations et des militants a conduit à l'instauration, à Paris, mais aussi dans d'autres villes, d'une commémoration annuelle à laquelle le Président de la République s'est associé cette année.

Il y a donc eu depuis vingt-cinq ans un important travail historique et mémoriel. Faut-il aujourd'hui aller plus loin, comme nous y invitent les auteurs de la proposition de loi ? Nous ne le pensons pas, et ce même si la formulation retenue par l'article 1 pour qualifier les événements du 17 octobre 1961, qui parle de « répression », ne fait pas polémique.

Il paraît impossible d'isoler le 17 octobre 1961 de son contexte et des violences liées à la guerre d'Algérie, violences qui ont touché toutes les communautés, y compris les Français musulmans d'Algérie, soumis à l'impôt révolutionnaire, à la guerre entre mouvements indépendantistes et à la pression policière. Je rappelle que cette dénomination administrative, « Français musulmans d'Algérie », résultait du choix fait par ceux-ci de se voir applique le droit local musulman plutôt que le code civil. À l'inverse, les personnes de confession juive des trois départements français d'Algérie- le Constantinois, l'Oranais, l'Algérois -ont accédé à la pleine citoyenneté en acceptant l'application code civil en 1870, par le décret Crémieux. Les réformes de 1944 et de 1956 avaient accordé à tous les citoyens vivant dans les trois départements d'Algérie les mêmes droits politiques et la citoyenneté complète. Il n'y avait donc plus de statut d'indigénat. La proposition de loi désigne les manifestants comme Algériens, ce qui, je le répète, est juridiquement inexact, mais j'ai pu constater que cette dénomination fait consensus chez les historiens. Plus complexe est le choix retenu par les auteurs de la proposition de loi de ne mentionner que la volonté d'indépendance comme motif de la manifestation. Une partie au moins des porteurs de mémoire du 17 octobre 1961 considère que la manifestation avait d'abord pour but de protester contre le couvre-feu de fait instauré par la préfecture de police.

L'article 2 a pour objet la création d'une commémoration annuelle. Les commémorations ont pour but de reconnaître la souffrance des victimes, que personne ne conteste ou ne minimise. Toutefois, reconnaître par la loi une commémoration suppose de reconnaître également les commémorations de toutes les autres victimes. Or il existe déjà une date, le 19 mars, qui à titre personnel ne me satisfait pas du tout, mais qui a été reconnue par la loi en 2012, et qui commémore toutes les victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. Par ailleurs, c'est par décret qu'ont été fixées la date du 25 septembre commémorant les forces supplétives de l'armée française, les harkis, et celle du 5 décembre pour la commémoration des morts pour la France pendant la guerre d'Algérie.

à l'occasion des soixante ans des événements tragiques du 17 octobre 1961. En présence de familles, de représentants et descendants de toutes les parties prenantes, il a observé une minute de silence en mémoire des victimes. Cette tragédie a longtemps été tue. Des cérémonies avaient été organisées par le maire de Paris ainsi que par d'autres élus de la Nation. La violence de la répression contre les manifestants du 17 octobre 1961 ne fait à présent aucun doute. Elle a été reconnue tant par le Sénat que par le Président de la République au travers de cette démarche. Par cet acte fort et courageux, c'est la première fois qu'un chef de l'État rend hommage aux victimes de la répression brutale, sanglante, du 17 octobre. Il a ainsi honoré leur mémoire en reconnaissant les crimes inexcusables pour la République commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon. Cela s'inscrit dans la démarche de lucidité engagée par le Président de la République sur toutes les blessures de l'histoire franco-algérienne. L'enjeu est en effet d'abord mémoriel, le travail historique devant se poursuivre. Le Président de la République avait confié à cet effet à Benjamin Stora un rapport sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. La commémoration de la répression du 17 octobre 1961 fait partie de la mise en oeuvre concrète des recommandations de ce rapport. Le Président de la République a déjà accompli plusieurs gestes de reconnaissance portant sur la période de la colonisation, avec la remise de restes humains à l'Algérie à l'été 2020, et sur celle de la guerre d'Algérie, s'agissant des assassinats de Maurice Audin et Ali Boumendjel, avec une plus grande ouverture de nos archives. Sur cette base, nous voulons que le dialogue puisse prévaloir avec nos partenaires algériens. Ce travail prendra du temps. Il passera par l'établissement des faits, par le dialogue des mémoires et par la mise en place patiente d'une relation apaisée avec notre passé commun. La proposition de loi que nous examinons ce jour est à plusieurs égards peu consensuelle- et pour cause ! Elle cherche à imposer une version de notre histoire, alors même que les historiens poursuivent un travail de fond. Comme je l'ai indiqué, le Président de la République a, avec courage, ouvert une voie par le dialogue et par des actes forts. Le Gouvernement souhaite que cette démarche se poursuive dans un esprit d'ouverture

il y a soixante ans, le 17 octobre 1961, à l'appel de la fédération de France du Front de libération nationale, au moins 20 000 Algériens ont défilé à Paris pour défendre pacifiquement une « Algérie algérienne » et dénoncer un couvre-feu imposé à ces seuls « Français musulmans d'Algérie ». Je crois qu'il n'y a aujourd'hui plus aucune ambiguïté quant au déroulement de cette manifestation et à l'ampleur de la violence qu'elle engendra alors de la part des forces de l'ordre. Le nombre de morts n'est pas exactement connu, mais, quelle que soit l'estimation, il est toujours édifiant. Au-delà du drame

dont les sociétés se racontent, voire se romancent à travers le temps. C'est un sujet évidemment difficile que celui de la question de la mémoire collective, du récit des événements que les générations offrent aux suivantes, les faisant

L'histoire est l'objet de discours et d'analyses à partir de recherches factuelles, de mises en perspective et de controverses parfois. Le passé n'a d'intérêt que parce qu'il est complexe, fait de sinuosités et d'enchevêtrements. Pour toutes ces raisons, la loi ne m'apparaît pas comme un support adéquat. Le fait historique ne s'écrit pas dans une sentence enfermée dans un article. J'y vois même un exercice périlleux

À cela s'ajoute ce que nous rappelons, hélas, trop souvent dans cet hémicycle : l'inflation législative. Nos lois manquent trop souvent d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire à l'essence de la fonction législative qui, pour citer Jean-Jacques Rousseau, devrait être de « découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux nations Une loi doit rester l'expression de la volonté générale dans l'organisation de la vie commune. Sa fonction n'est pas de livrer une analyse historique, aussi juste soit-elle. Laissons ce travail aux historiens Les livres, les revues et les encyclopédies qu'ils écrivent sont destinés à mettre en lumière le rôle de chacun dans les événements, à reconstituer et décrire des faits avec le souci du détail.

dans la répression de manifestants algériens réclamant pacifiquement l'indépendance de leur pays ayant eu lieu le 17 octobre 1961 et les jours suivants à Paris ». Eh bien, voilà ! Je crois que cette démarche a été amorcée depuis longtemps. Sur la forme, une loi n'est pas le support qui permet de dresser un tel constat : un événement historique ne saurait être réduit à la simplicité d'une phrase.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la gauche nous propose de voter un texte de loi reconnaissant la responsabilité de la France lors de la manifestation des militants du FLN du 17 octobre 1961, une gauche qui porte aujourd'hui cette proposition de loi, comme elle portait les valises autrefois, motivée par la haine de la France. Petit rappel des faits et uniquement des faits. Le 17 octobre 1961, le FLN, mouvement terroriste se réclamant du socialisme, qui a assassiné plus de 6 000 Algériens en métropole entre 1955 et 1962, qui a commis des actes abominables envers les civils français et les harkis dans nos départements en Algérie, ce ramassis d'assassins appelle donc à manifester en plein coeur de Paris. 20 000 soutiens à un mouvement terroriste manifestent et provoquent la police qui ne fait que rétablir l'ordre. Quelques jours après, la propagande du FLN et le parti communiste français, jamais en retard d'une collaboration avec l'ennemi ni d'un mensonge historique, ... Et les résistants allant jusqu'à évoquer des centaines de morts du côté du FLN. Cette propagande anti-française se heurte à une réalité, mes chers collègues : un seul cadavre a été ramené à l'institut médico-légal de Paris ce soir-là, celui de Guy Chevalier, tué lors de la manifestation. Jean Géronimi,

1961. Quand la justice ne donne pas raison à la gauche, celle-ci n'hésite pas à redoubler d'exagérations, de mensonges et de manipulations pour tenter de faire condamner la France. vous êtes des faussaires de l'Histoire, car vous oubliez sciemment tous les Européens, nos compatriotes pieds-noirs et harkis, ... Ah ! ... « compris », puis trahis par le général élyséen et massacrés par les barbares du FLN, comme à Oran le 5 juillet 1962. Ces victimes-là sont peut-être trop françaises pour mériter votre compassion ... Si vous aviez un peu d'honnêteté historique et politique, vous demanderiez au gouvernement algérien d'ouvrir ses archives ; et, après que la vérité a éclaté, vous exigeriez que l'Algérie présente ses excuses aux familles des victimes et à la France. Allez jusqu'au bout ! Vous voulez la vérité ? La voilà : les pieds-noirs, ces Français, ont accompli une oeuvre extraordinaire sur cette terre française qu'était l'Algérie. La France a créé l'Algérie, le FLN l'a ruinée C'est si vrai que des millions d'Algériens, pourtant riches d'une patrie, ont préféré la fuir pour trouver refuge dans l'ancien pays prétendument colonisateur, réellement civilisateur, ... Voilà l'extrême droite ! ... et qu'ils sont encore des millions à vouloir trouver en France un espoir d'avenir. Hier, la gauche trahissait la France ; aujourd'hui elle veut déconstruire et falsifier son histoire. Nous ne vous laisserons pas faire ! Je ne vous laisserai pas salir une fois de plus la France et les Français ! Mes chers collègues, je vous invite à me rejoindre sur les barricades de la vérité, à « porter haut et fier ce beau drapeau de notre France entière » en rejetant cette proposition de loi

que dire après un tel discours,

soit, les historiens ont depuis longtemps produit un travail scientifique indiscutable sur cette journée du 17 octobre 1961. Ils ont établi les faits. Ils les ont inscrits dans les livres afin que rien ne les efface. Ils disent la mécanique à l'oeuvre durant plusieurs mois, tout au long de cette année 1961, à ce moment de notre histoire où les valeurs de la République ont été reléguées. Au premier rang de ces valeurs figure la liberté : celle d'être qui l'on est, sans jamais risquer d'être condamné pour ce celle de pouvoir exprimer son opinion et de la défendre dans le débat public ; celle de manifester pacifiquement. Oui, avec lucidité, notre pays reconnaît que les actes commis sous l'autorité de Maurice Papon sont bien des crimes et qu'ils sont inexcusables pour la République. Ce n'est pas là une opinion : c'est un fait. Le souvenir du 17 octobre 1961 porte en lui une singularité. Il s'agit d'un processus de construction mémorielle populaire. Depuis des dizaines d'années, cette mémoire s'est construite par la volonté de nos concitoyens, par-delà les origines, les racines et les obédiences. La flamme de son souvenir a été allumée et entretenue. Elle ne s'éteindra pas. Cette mémoire est vivante.

Il ne s'agit pas de créer une journée nationale supplémentaire. Je le répète, cette proposition de loi est une étape dans un processus au long cours. Il y eut d'abord la pose d'une plaque commémorative, le 17 octobre 2001, par Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, puis la reconnaissance lucide du président François Hollande, le 17 octobre 2012. Entre 2012 et 2017, mon prédécesseur et moi-même, en qualité de secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, avons oeuvré au rassemblement de toutes les mémoires en nous appuyant sur la science des historiens. Ainsi, j'ai longuement travaillé avec des scientifiques de toutes les sensibilités historiographiques, notamment avec le professeur Jim House, spécialiste incontournable

d'un long et lent processus. C'est le sens de la mémoire, cette chaîne dont chaque citoyen est un maillon ; cette chaîne qui nous vient du passé et tend vers l'avenir. La France est un grand pays. Cela ne l'immunise pas au regard de l'histoire. Cela ne l'exonère pas non plus. La France est un grand pays, justement parce qu'elle est capable de regarder son passé avec discernement, d'en connaître les événements, de se réjouir de toutes les fois où elle a été à la hauteur, de reconnaître aussi les moments où elle n'a pas su s'élever. Par son esprit de résilience, la France est digne pour tous ceux qui la regardent et lui font confiance. J'en ai mesuré la force lorsque, en avril 2015, je me suis rendu à Sétif, en Algérie.

L'humanité, lorsqu'elle est ainsi frappée, n'a plus de nationalité. Il ne reste que des mémoires douloureuses, qui toutes doivent être honorées. J'ai, une nouvelle fois, mesuré la force de la réconciliation des mémoires lorsque, en janvier 2016, je me suis rendu devant la plaque commémorative du pont Saint-Michel afin d'y déposer une gerbe avec mon homologue algérien, Tayeb Zitouni, ministre des moudjahidines. En ces instants, notre pays a mis en adéquation ses valeurs et ses actes, sans avoir peur d'effectuer un travail d'analyse.

celle du bourdonnement incessant des magazines et des journaux, des réseaux sociaux et des chaînes de télévision. Une certaine mode voudrait que notre pays décline. La science, le travail patient des historiens, la vérité des faits, tout cela lui est étranger. Cette mode permet à certains de vendre et de bien vivre, puisqu'ils en font monnaie. Prenons garde ! Si ces peintres de mauvaise facture venaient à prendre le pouvoir, ils représenteraient un danger pour la démocratie. Ce texte est l'un des éléments- pas le seul -permettant aux générations actuelles et futures d'avancer sans peur ni reproche. C'est un pas supplémentaire vers la concorde mémorielle. Notre pays suit ce chemin sans rien oublier des violences, où qu'elles aient frappé ; en pensant à tous les déracinés, à tous ces enfants, ces femmes et ces hommes qui ont dû abandonner une vie entière en quelques heures

Dans le respect de la mémoire de toutes les victimes, françaises et algériennes, je tiens à le dire clairement : la France fait son travail de mémoire. Elle le prouve encore aujourd'hui. Mais elle ne peut pas le faire seule. L'apaisement des mémoires appelle chaque pays à oeuvrer dans ce sens et à s'en donner tous les moyens. Continuons donc d'avancer ensemble

algériens le 17 octobre 1961, dans le contexte très violent de la guerre d'Algérie. Le présent texte traite de ce sujet deux objets distincts : d'une part, l'inscription dans la loi de la responsabilité de la France dans cette répression d'autre part, l'inscription dans la loi de la commémoration de ces événements, chaque 17 octobre. Sur le second point, il n'est pas inutile de rappeler qu'une commémoration peut être célébrée sans qu'intervienne une loi. le Président de la République a participé à la commémoration de cette répression en octobre dernier, en présence de descendants des différents porteurs de mémoire.

Nous ne sommes pas de ceux qui ont regretté ce geste en lui opposant d'autres mémoires : l'objectif était justement de les convoquer ensemble autour du drame du 17 octobre 1961.

il risque d'entraîner dans la mémoire une parcellisation des drames, y compris au sujet des derniers mois de la guerre d'Algérie. Ce risque nous rappelle bien la nécessité du travail d'association et de décloisonnement des mémoires, dont l'objectif de pacification pourra susciter un consensus assez large sur ces travées. La commémoration précitée, à laquelle le Président de la République, Emmanuel Macron, a procédé le 16 octobre dernier ; sa reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la mort du mathématicien Maurice Audin et des tortures qu'il a subies, ainsi que de l'assassinat de l'avocat et nationaliste algérien Ali Boumendjel ; la démarche de facilitation de l'accès aux archives ; ou encore

République. Il a exprimé sa volonté d'entendre « un grand discours sur la guerre d'Algérie, qui reflète toutes les mémoires : celle des indépendantistes, des juifs d'Algérie, des pieds-noirs, des harkis, des appelés. Un discours qui ne se contente pas d'énumérer ces mémoires, mais au contraire les intègre dans un narratif d'ensemble, leur permette d'exister ensemble ». Faisant sienne cette volonté de dépassement et de décloisonnement, le groupe RDPI s'abstiendra. La parole

pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là et les jours suivants, nous devons nous souvenir de cette période sombre de notre histoire. En effet, 1961 est une année de troubles, la France étant alors en guerre depuis sept ans, la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie, colonisée depuis 1830, se poursuit. La question de cette indépendance divise profondément notre société.

cette même année 1961. Elle a fait plus d'un millier de morts tout au long de son existence. Son dirigeant, le général d'armée Raoul Salan,

Malgré ce climat de violence, le général de Gaulle se prononce en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Le 12 juillet 1961, il déclare : « La France accepte sans aucune réserve que les populations algériennes se constituent en un État entièrement indépendant. » En dépit de cette déclaration sans équivoque, les violences continuent. Des attentats sont perpétrés, notamment à l'encontre des policiers. Dans ce climat de forte tension, le préfet de police de Paris, Maurice Papon, impose aux seuls «

il importe de les replacer dans leur contexte. En 2012 et en 2018, les présidents de la République François Hollande, puis Emmanuel Macron, ont rendu hommage à la mémoire des victimes et ont reconnu la responsabilité de notre République. Plusieurs membres du groupe socialiste nous invitent aujourd'hui à voter une proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de la France dans la répression sanglante de cette manifestation. Il semble pourtant que deux présidents de la République ont déjà satisfait cette demande. Nos collègues proposent également d'organiser chaque 17 octobre une commémoration officielle rendant hommage aux victimes. Cette suggestion pose nécessairement question : pourquoi commémorer cet épisode plutôt que d'autres ? Cette guerre, comme toutes les guerres, ne manque, hélas ! pas d'événements tragiques. Faut-il les commémorer tous, au risque de banaliser les commémorations ? Nous en sommes persuadés : notre devoir est aujourd'hui de nous tourner vers l'avenir.

nul ne remet sérieusement en question la violence de la répression contre les manifestants du 17 octobre 1961. À cet égard, il n'y a aucun doute : cette réalité a été reconnue comme telle.

le président de la République déclarait : « Des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. » En octobre 2021, l'actuel chef de l'État ajoutait quant à lui : « Les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République. Rappelons d'ailleurs que cette déclaration s'inscrit dans la continuité des préconisations du rapport Stora, commandé en juillet 2020, sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Pour autant, la responsabilité de la France, telle que l'article 1 propose de la reconnaître, n'a pas fait consensus au sein de notre commission.

on reste surpris des intentions sous-jacentes de ce texte et des amendements déposés par ses auteurs, dont nous aurons à discuter. Ainsi, le terme de « crime d'État » que certains veulent retenir est non seulement impropre mais irresponsable, particulièrement quand on voit comment, de l'autre côté de la Méditerranée, le pouvoir militaire en place tronque et instrumentalise cet épisode tragique pour faire le procès de la France ; quand on constate l'existence d'une certaine rente mémorielle, que d'aucuns cherchent à alimenter, sans doute pour obtenir de notre pays un supplément de repentance et- pourquoi pas ? -une indemnisation. Par conséquent, telle qu'elle est présentée, la question de la responsabilité de la France paraît trop générale, générale, à ceux qui souhaitent l'assignation claire et nominative de responsabilités comme à ceux qui refusent de voir imputée à la Nation entière la responsabilité d'actes illégaux. C'est pourquoi notre commission des lois s'est, à raison, prononcée en défaveur de ce texte du groupe socialiste : selon elle, la reconnaissance et les commémorations prévues ne sont pas susceptibles de « contribuer à l'apaisement et au travail mémoriel commun ». Faut-il rappeler que le Président de la République lui-même évoquait les « sables mouvants de la mémoire »

Autrement dit, l'approche mémorielle demeure forcément délicate et malheureusement sujette à manipulations, compte tenu des circonstances historiques et d'un contexte caractérisé par les attentats du FLN en métropole. En vertu de l'article 1 du présent texte,

qu'elle devrait expier par des rituels collectifs de contrition et autres programmes de réparation symbolique, sous forme notamment de discrimination positive en direction de chaque boutique victimaire. Je suis de ceux qui refusent cette injonction à l'expiation. N'entrons pas dans l'engrenage des mémoires concurrentes, phénomène largement analysé par les historiens, qui nous mettent en garde contre les lois mémorielles depuis une vingtaine d'années. Méfions-nous-en d'autant plus que le travail historique relatif à la guerre d'Algérie a largement été réalisé et qu'il se poursuit.

du souvenir et de recueillement à la mémoire [de toutes les] victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ». Gardons-nous de confondre le travail des historiens et celui du législateur. Toutes les lois mémorielles ne sont pas les bienvenues ... Ah ! Il appartient aux historiens, dont c'est le domaine de compétence, de rappeler ce que la France a fait et n'a pas fait.

présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestent pour le droit à l'indépendance sont tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits », a déclaré François Hollande en 2012, avant qu'un autre président de la République, Emmanuel Macron, n'ajoute : « Les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République. La France regarde toute son histoire avec lucidité et reconnaît les responsabilités clairement établies. Ces deux déclarations s'inscrivent dans un travail de mémoire, un travail académique pour dire la vérité historique et établir la responsabilité de l'État. Il s'agit d'un mouvement qui part de la connaissance pour aller vers la reconnaissance. Ce travail, entamé depuis des années, a été renforcé par l'approche retenue par Benjamin Stora dans son rapport du début 2021.

mais recommande des avancées sur des chantiers pragmatiques, une politique des petits pas supposant, par exemple, l'ouverture des archives et la reconnaissance du 17 octobre comme un crime d'État.

Yannick Jadot l'a rappelé : « Le Président a raté l'occasion de faire un pas de plus vers la réconciliation. » Et ce n'est pas le seul à avoir gâché une occasion d'apaisement. En témoigne la position de notre rapporteure, qui, dans cette proposition de loi, voit au mieux une reconnaissance redondante de la violence de la répression contre les manifestations

un argument byzantin, certains veulent à tout prix différencier la responsabilité de la France de celle du préfet de police de la République. Les événements du 17 octobre 1961 ne sont pas ponctuels ou inopinés.

Qu'il y ait d'autres coupables ne fait pas de vous un innocent ! D'autres estiment que cette reconnaissance irait à l'encontre d'un objectif d'apaisement. Pour leur répondre, je ne saurais trop leur répéter cette citation, souvent attribuée à ce fils d'Algérie, Marseillais d'adoption, Albert Camus : « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je n'ose croire que votre croyance forte en un « parler vrai », en d'autres termes dire la vérité même quand elle dérange, atteindrait ses limites lorsqu'il s'agit de notre histoire. Benjamin Stora, l'un des historiens au coeur de cette réflexion, s'est prononcé contre l'idée d'excuses officielles.

le sujet est sensible et complexe. Le conflit en Algérie était bien une guerre. Elle a laissé des cicatrices profondes, y compris chez les pieds-noirs et chez les juifs pieds-noirs, dont je fais partie.

Après des années de silence officiel, de déni et d'occultation, la mémoire militante de la dénonciation commençait enfin à s'exprimer, presque sans crainte. Le 17 octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie, des Algériens manifestent pacifiquement à Paris contre le couvre-feu discriminatoire décrété par le préfet de police Maurice Papon, lequel était imposé à tous les Algériens vivant en région parisienne.

sans compter les nombreux blessés et les 11 000 arrestations qui suivirent dans des centres de détention spécialement mis en place. De la mémoire des faits à leur reconnaissance officielle, plusieurs années se sont encore écoulées jusqu'au communiqué de presse de François Hollande en 2012, cinquante ans après le massacre ! La même année, le groupe communiste du Sénat

Plus récemment, en juillet 2020, souhaitant « réconcilier les mémoires autour de la colonisation et la guerre en Algérie », Emmanuel Macron demandait un rapport en ce sens à l'un des historiens spécialistes du sujet, Benjamin Stora. Les auteurs de la présente proposition de loi s'appuient en grande partie sur le contenu de ce rapport remis au début de l'année, qui préconise « la poursuite de commémorations », notamment pour ce qui concerne la « répression de travailleurs algériens en France

Comme le rappelait déjà notre groupe en 2012, ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 n'était pas un événement isolé survenu en un lieu et en un moment unique. Cela constitua le paroxysme d'une politique de guerre coloniale symbolisée par la mise en place du sinistre préfet de police Maurice Papon.

D'autres dates nous rappellent à quel point la violence d'État fut indissociable du colonialisme : la répression du 8 mai 1945 à Sétif, les massacres de Madagascar en 1947, la terrible guerre d'Indochine, la torture pendant la guerre d'Algérie, la funeste bataille d'Alger, la « disparition » du mathématicien Maurice Audin et le massacre du 8 février 1962 au métro Charonne en furent des épisodes particulièrement violents. La mémoire lucide et apaisée sur ces événements n'existe pas encore. C'est la raison pour laquelle nous devons adopter cette proposition de loi. Enfin, nous considérons pour notre part qu'il serait nécessaire d'ouvrir les archives sur le sujet, notamment celles de la police et de la justice, et, au-delà, toutes les archives relatives aux guerres coloniales et à leur cortège de répression et de massacres. Ces dispositions compléteraient utilement celles proposées aujourd'hui, qui recueillent tout notre soutien.

une commémoration officielle leur rendant hommage. Le groupe Union Centriste n'y souscrit pas. Notre rapporteure, dont nous partageons les conclusions et dont je salue la pondération et l'objectivité, a montré que l'idée d'une responsabilité générale de la France n'était pas pertinente. En effet, les actes atroces, illégaux, commis à l'encontre des manifestants ont été perpétrés sous l'autorité du préfet de police et de ses complices, et non par la Nation tout entière. la rapporteure a rappelé le dissensus historique quant aux motivations des participants, qui manifestaient soit pour l'indépendance de l'Algérie, soit contre le couvre-feu imposé aux Français musulmans d'Algérie. Ce point fait s'interroger sur la consécration législative de cette seule date, à l'exclusion de tant d'autres tout aussi tragiques et douloureuses.

après que tant de policiers ont été tués. Je vous livrerai quelques interrogations, sans prétendre à l'exhaustivité. L'apaisement mémoriel doit-il être recherché ? Oui, bien sûr,

les massacrés à Oran le 5 juillet 1962, pour ceux qui vivent ou portent en héritage l'affliction de la confiance trahie : certains s'en remettaient à la parole de la France, d'autres aux engagements du FLN, d'autres encore ont cru au respect des accords d'Évian. L'apaisement mémoriel doit être également recherché pour les ouvriers des grands chantiers routiers du plan de Constantine qui ont été assassinés, mais aussi pour les professeurs exécutés, et pour les 27 817 jeunes Français mobilisés ou engagés qui ne sont pas revenus d'Algérie pour les 1 630 Européens enlevés par le FLN et disparus, pour les supplétifs, les harkis, les moghaznis ; pour les 150 000 personnes abandonnées à la vengeance comme pour les 40 000 ramenées en France, rarement avec leurs familles et dans quelles conditions, sans aucune considération ;

pour ces jeunes lieutenants qui, soixante ans après, se demandent encore s'ils ont bien fait, conformément aux ordres, d'inciter leurs tirailleurs à rejoindre les forces locales de libération avant, dans bien des cas, d'apprendre leur exécution

pour les proches et les descendants de tous ceux-là, pour les descendants de juifs et d'occidentaux inhumés en Algérie dans des cimetières dont l'entretien est inexistant. Pour eux aussi, nous devons travailler à l'apaisement mémoriel

Le groupe « Regards de la jeune génération sur les mémoires franco-algériennes », qui réunit les petits-enfants de chaque camp autour du Président de la République, a des réponses plus subtiles, plus globales, moins partielles, peut-être aussi moins partiales. Ce texte contribue-t-il à la réconciliation et au renforcement de nos liens avec l'Algérie ? Je ne le pense pas davantage. La repentance unilatérale n'a pas conduit à un apaisement partagé, bien au contraire. Quels pas l'Algérie a-t-elle esquissé après la commémoration du 17 octobre présidée en 2012 par le président Hollande ? Après la loi du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ?

L'État algérien, enfermé dans le dogme d'une histoire officielle et d'une « rente mémorielle », pour reprendre les mots justes que le Président de la République a prononcés au mois de novembre dernier, n'a fait aucun pas. Il s'indigne, il insulte, il instrumentalise. L'apaisement mémoriel ne peut être unilatéral et partiel. Les auteurs de la proposition de loi proposent que ce soit la France tout entière qui regarde avec lucidité son histoire, toute son histoire. l'apaisement mémoriel n'est envisageable que si la France tout entière et l'Algérie tout entière regardent ensemble avec lucidité, vérité et justice leur histoire commune, toute leur histoire commune.

aux victimes de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, est avant tout une démarche idéologique et politicienne. Une fois de plus, cette initiative malvenue se détache totalement du contexte difficile de l'époque pour verser, encore et toujours, dans l'autoflagellation mémorielle.

et qui, hasard du calendrier électoral, change de position et appelle finalement hier à ne pas la revoir. Pourquoi vouloir également commémorer cette date et aller aussi loin en reconnaissant la responsabilité de la France ? Les célébrations du 19 mars, que la gauche a imposées par une manoeuvre grossière, ne vous suffisent-elles

terrible période. Oui, nous étions en guerre, et ce tragique épisode s'inscrit dans un temps douloureux de l'histoire. Oui, la guerre était en Algérie, mais elle était aussi en métropole. La métropole n'était pas en guerre ! Oui, l'organisation terroriste du FLN a tué et massacré des soldats

Bravo ! Ne vous en déplaise, l'Histoire est bien plus complexe que vous ne l'écrivez. Il faut bien plus que deux lignes dans une proposition de loi pour en rendre compte. compte. On ne peut pas discuter de cette proposition de loi si l'on continue à sélectionner les mémoires et à rejeter certaines douleurs, comme le massacre « oublié » d'Oran du 5 juillet 1962.

Le ministre des affaires étrangères Le Drian devrait avoir le courage de le rappeler aux autorités algériennes lors de sa visite aujourd'hui ... Cette proposition de loi consacre encore inutilement la concurrence des mémoires, au détriment de ceux qui ont choisi la France. Arrêtons de prétendre que seule la France aurait commis des fautes durant cette guerre ! On ne peut pas exonérer le FLN et ses complices porteurs de valises de leurs responsabilités. On ne peut pas rendre la police, que vous visez sans la nommer, comme la seule et unique responsable de ce cycle de violence tragique. Ce sens unique mémoriel que vous consacrez dans cette proposition de loi est insupportable. Insupportable, car ce texte alimente la propagande victimaire anti-France ... Bravo ! ... et érige les victimes des affrontements en martyrs de la cause algérienne. Insupportable, car il étaye le communautarisme et le séparatisme.

Depuis des décennies, ceux qui ont vécu cette douloureuse histoire sont instrumentalisés par les gouvernements français et algérien. Les pieds-noirs et les harkis en ont assez. Ils veulent vivre- et malheureusement, pour certains, mourir -en paix, loin de leur terre natale, et ne plus avoir à supporter ces attaques permanentes contre ce qu'ils étaient. Albert Camus écrivait que les gens de sa famille n'avaient « jamais exploité ni opprimé personne ». Laissons le passé aux historiens et cessons de vouloir le réécrire à grand renfort de lois dont l'objectif est avant tout de s'attacher les bonnes grâces d'une partie de l'électorat.

Je connais ces déchirements mieux que vous. Certains y ont laissé la vie. D'autres ont tout perdu, y compris leurs racines. La politique de réparation ne peut se résumer à l'expiation permanente par la repentance, qui aboutit à la division. La France est une nation qui revendique son identité et qui assume son histoire. Mais comme n'importe quel autre pays au monde, elle peut reconnaître ses torts et réserver ses célébrations pour ses heures les plus glorieuses. Non, il n'y a rien à célébrer le 17 octobre, pas plus que le 19 mars. Ce sont des dates de sinistre mémoire qui riment avec peine et douleur. Pour conclure, je suis persuadé que les Français ont besoin de croire en la France.

Nous souhaitons, pour notre part, montrer à nos enfants et à tous nos concitoyens qu'il existe encore pour eux et pour la France un autre chemin que celui de la résignation. Un chemin qui conduit à la grandeur de notre pays et qui respecte son histoire. La France doit se rassembler autour d'une espérance, celle d'un tout, et non d'une addition choisie de morceaux de l'Histoire, surtout lorsque ces derniers ne servent qu'une fin : une logique victimaire au mépris de ceux qui ont choisi la France pour ce qu'elle était et pour les valeurs qu'elle portait. Pensons à eux en cet instant et honorons-les pour avoir fait en toutes circonstances un seul choix : celui de la France.

dont certaines avaient fait l'objet d'une déclaration à la police. Ces mêmes historiens ont établi ces faits de longue date et les ont resitués dans un engrenage de violences qui, en fait, a duré plusieurs semaines.

La question de la contextualisation des événements du 17 octobre 1961 est importante. Tous les orateurs l'ont souligné dans leurs interventions. Cependant, cet amendement pose un problème de contexte : l'article 1 vise la répression de la manifestation du 17 octobre en tant qu'événement singulier.

à imposer une certaine version de l'histoire officielle. Le travail des historiens appartient aux seuls historiens, et ce travail est en cours. Nous faisons confiance à ces professionnels des sciences humaines pour nous éclairer sur les faits. Le Gouvernement est donc défavorable

M. Guy Benarroche. La dénonciation par Emmanuel Macron de « crimes inexcusables pour la République » est une première pierre à l'édifice de la reconnaissance officielle de ce massacre. Cette déclaration ne va cependant pas assez loin. Tout d'abord, nous considérons que, bien que la répression ait été orchestrée par le préfet de police de Paris, Maurice Papon, la responsabilité de tels massacres est à chercher au plus haut sommet de l'État français et qu'elle découle à la fois d'une décision et d'un contexte politique.

Enfin, les travaux des historiens montrent que la violence de la répression du 17 octobre 1961 est à mettre en regard des techniques de répression coloniale : près de 12 000 Algériens furent arrêtés et transférés dans des centres de tri, au stade de Coubertin et au palais des sports notamment. Certains furent torturés lors de leur interrogatoire par les forces de l'ordre. Dans un souci de retranscription de la vérité et de transmission de la mémoire, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande à ce que soit reconnue comme crime d'État la répression sanglante des manifestants algériens qui a été commise sous l'autorité du préfet de police de Paris Maurice Papon.

Le scrutin est ouvert.

les années sombres de la guerre d'Algérie, y compris la répression du 17 octobre 1961 et les jours qui la suivent. Cette promesse a rapidement été rompue par le Gouvernement lui-même qui, profitant de la loi Sécurité globale,

Au-delà de cette restriction, je pense aux familles qui vivent dans la douleur et l'incompréhension de leur propre histoire. Longtemps, il a existé une omerta sur cette partie de l'histoire franco-algérienne.

puisque celle-ci se trouve dans les archives, dont une part seulement est accessible. Il est temps, soixante ans après, de soigner cette blessure mémorielle. Il est de notre devoir de contribuer à ce travail d'histoire et de mémoire, en ouvrant définitivement l'accès aux archives à tous les citoyens, afin de compléter les travaux historiques déjà engagés. Le droit à l'information, à la recherche, à la science est inaliénable.

Je rappelle aussi que M. Jean-Paul Brunet a écrit deux ouvrages sur le sujet, qui reposent sur une exploitation particulièrement minutieuse

Quel est l'avis du Gouvernement ?

sur ce sujet, qui est très important.

Monsieur Bonhomme,

j'ai bien noté que chacun était d'accord pour admettre les faits. Chacun reconnaît qu'il y a eu une terrible répression, avec des centaines de blessés et des morts parmi les personnes arrêtées par les forces de police.

Nous souhaitons tous normaliser les rapports avec l'Algérie. Mais l'apaisement et la réconciliation ne peuvent prendre corps que sur le socle de la réciprocité. C'est pourquoi je ne voterai pas cette loi.

cette date, qui n'est pas une date ordinaire. Elle a donné lieu à un drame absolument épouvantable dans les rues de Paris- et si nous ne savons pas tout, au moins connaissons-nous l'ampleur de l'horreur de cet événement. Voilà ce qu'il s'agit de renforcer

il appartient au président de séance d'appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ». L'expression « il appartient au président de séance » montre certaine marge de manoeuvre. Par ailleurs, dans la formation que vous souhaitez avoir sur les pratiques et les moeurs du Sénat, je vous suggère d'inclure une formation au sens de l'humour.

incongrues et partisanes. Jusqu'à présent, personne n'avait jamais mis en cause ni ma présidence ni celle de mes collègues vice-présidents.

Il ne s'agit pas de faire un concours entre différentes mémoires sur d'autres événements tragiques, que vous avez rappelées et que je partage. Il ne s'agit pas non plus de faire un concours avec le gouvernement algérien pour savoir si c'est lui qui doit faire le premier pas, ou notre

Au-delà du constat, si l'on cherche à comprendre les mécanismes en jeu, on mesure à quel point le rapport à la politique a changé. Il a changé par les combats que les jeunes portent féminisme, cause animale, écologie, droits des LGBT. Mais aussi par la manière de les mener ; la politique passe moins par les partis que par les réseaux sociaux, davantage par la manifestation ou la pétition que par le vote. Mais oui, la jeunesse est politisée, concernée, en attente et exigeante. Elle est présente dans la vie associative, la démocratie scolaire et participative, et le désir d'engagement progresse chez les jeunes. Il convient cependant d'ajouter à la réflexion qu'il y a des jeunesses, qui ont des rapports différents à l'engagement et à la politique. Mais on ne peut en rester là, se résigner à voir chaque soir d'élection l'abstention augmenter de manière structurelle. On ne peut passer plus longtemps à côté de la possibilité de faire d'une génération engagée une génération citoyenne. On ne peut passer plus longtemps à côté de la possibilité de faire d'une démocratie « sans citoyens », qui conçoit les jeunes comme une catégorie qu'il faut tenir à distance, une démocratie partagée. reprendre les propos de Léon Blum : « Toute classe dirigeante [qui n'est pas capable] d'employer la force fraîche des générations montantes, est condamnée à disparaître de l'histoire. On mesure alors que si rien n'est fait pour prendre en compte les jeunes et les valeurs qu'ils portent, nous courrons le risque qu'ils disparaissent du champ politique et fassent définitivement sécession, selon l'expression de Frédéric Dabi dans son ouvrage. Il est Il est donc temps de leur tendre la main, de leur adresser un message fort de confiance et de responsabilisation, de leur dire que nous voulons faire République avec eux. La proposition de loi présentée aujourd'hui traduit cette urgente nécessité. Elle prévoit d'abaisser l'âge du vote à 16 ans avec une « préparation » par l'introduction d'un enseignement évalué de sciences politiques au collège, en renforcement de l'éducation morale et civique, une formation spécifique des enseignants et la généralisation des conseils municipaux de jeunes dans les communes de plus de 5 000 habitants et les départements, avec un nombre minimal de jeunes. Cette proposition d'abaissement de l'âge du vote se veut une réponse, certes parmi beaucoup d'autres, à l'abstention. Elle s'appuie sur les travaux de nombreux chercheurs, dont ceux d'Anne Muxel, sociologue et directrice de recherche au Centre de l'habitude de voter est prise de façon précoce, plus on a de chances de devenir un électeur systématique dans le cours ultérieur de sa vie. Elle souligne notamment qu'il suffit qu'une personne ait voté trois fois dans la foulée de son entrée dans la citoyenneté active pour que les chances de la voir participer ultérieurement soient fortes. À 16 ans, la famille et l'école jouent un rôle de cadre favorisant la pratique du vote. Au contraire, 18 ans est l'âge de la décohabitation familiale, propice à la « mal-inscription », l'âge de la recherche de son avenir professionnel, universitaire et sentimental. Pourquoi 16 ans ? À cet âge, la société accorde déjà de nombreux droits, tendant à prouver que l'on est mûr, responsable à ce stade. Ainsi, tout mineur peut être émancipé une fois l'âge de 16 ans atteint, travailler, consentir à l'impôt, s'immatriculer à la sécurité sociale, reconnaître un enfant, obtenir un permis de chasse, faire un testament, effectuer un service civique, choisir son médecin, être pompier volontaire, créer une association, etc. En un mot, on est considéré comme adulte ! Alors, comment expliquer que l'on ne puisse exercer un droit de vote pour peser sur les décisions qui vont impacter son avenir ? Plusieurs États ou pays dans le monde et en Europe ont rendu effective la majorité élective à 16 ans pour les élections locales et/ou nationales, à certaines conditions ou non, et d'autres s'apprêtent à le faire, comme l'Allemagne. Le Conseil européen, dès 2015, recommande dans une résolution d'envisager d'harmoniser l'âge minimal des électeurs à 16 ans afin de garantir aux citoyens de l'Union une plus grande égalité lors des élections.

Ce mouvement s'inscrirait dans le sens du progrès, du renforcement de la démocratie et dans la longue histoire de la conquête du droit de vote, du suffrage universel au vote des femmes, jusqu'à l'abaissement de la majorité électorale à 18 ans. Voter à 16 ans, c'est le cours de l'Histoire. Il faut prendre acte du caractère de plus en plus précoce de l'autonomie des jeunes. Certes, ils restent dépendants financièrement des parents plus longtemps, mais ils sont aujourd'hui plus que jamais capables d'autonomie dans leurs contacts et leurs modes de socialisation, car plus mobiles, plus informés, plus formés. Ils pourraient ainsi peser sur les décisions politiques qui les concernent. Mais pour que ce droit soit pleinement efficace, il faut permettre à tous de construire une réflexion politique libre et éclairée. L'école, « fabrique des citoyens », est la plus à même de donner les clés de compréhension de la société, de développer l'appétit à la vie de la cité, aux idées politiques, à la philosophie et à l'histoire politique. C'est pourquoi l'article 2 de la proposition de loi prévoit la création au collège d'un enseignement en sciences politiques dont les savoirs spécifiques permettront d'édifier la citoyenneté, en complément de l'enseignement civique et moral, et avec des méthodes adaptées. L'article 3 prévoit la généralisation des conseils de jeunes dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les départements. À côté de l'école, de la famille, des associations, les jeunes aspirent à s'exprimer localement sur des thématiques qui touchent au vivre-ensemble, aux solidarités, à l'intergénérationnel, à l'environnement. C'est une manière d'offrir à des dizaines de milliers de jeunes l'opportunité d'être partie prenante de la démocratie locale et de s'initier au fonctionnement d'une collectivité territoriale. Il s'agit d'un dispositif essentiel, actuellement sous-utilisé, qui peut contribuer à la construction d'un parcours citoyen complet des jeunes. Face aux multiples crises que nous affrontons- sanitaire, écologique, démocratique deux attitudes sont possibles. On peut se renfermer sur soi-même, frileusement, en cultivant la peur et le rejet de l'autre. La jeunesse est alors une menace, une turbulence qu'il faut contenir, contrôler et tenir à distance. l'on peut, comme nous vous le proposons, envisager un avenir ouvert, enthousiaste, optimiste et généreux qui croit aux générations futures, celles qui feront le monde de demain. La jeunesse est alors une ressource, un interlocuteur politique compétent et légitime. Notre pays ne peut rester immobile, notre démocratie est fatiguée. Donnons-lui un nouveau souffle en faisant confiance aux jeunesses, car elles nous attendent et elles le méritent.

Cette proposition de loi part d'un constat, malheureusement renouvelé élection après élection, celui de l'abstention massive des jeunes âgés de 18 à 36 ans aux élections politiques. Afin d'y remédier, elle met en avant deux instruments l'ouverture du droit de vote dès l'âge de 16 ans, d'une part, et l'institution de conseils de jeunes dans toutes les communes de plus 5 000 habitants ainsi que pour les conseils départementaux, d'autre part. Elle vise également à accompagner l'abaissement de la majorité électorale en prévoyant un nouvel enseignement obligatoire en sciences politiques et en histoire de la vie politique française et européenne pour les élèves de collège. La formation des enseignants serait également adaptée en conséquence. L'article 1, qui vise à abaisser la majorité électorale à 16 ans, constitue la mesure phare du texte, qui n'a pas convaincu la commission. Nous ne pouvons évidemment qu'être d'accord avec la nécessité de lutter contre l'abstention des jeunes ; pour mémoire, la participation aux élections régionales et départementales de 2021 s'est élevée à seulement 17 % chez les 18-24 ans, et

Pour autant, la solution proposée, à savoir ouvrir le droit de vote à une nouvelle tranche d'âge plus jeune, ne nous semble pas opportune pour des raisons à la fois de principe, juridiques et sociologiques. Tout d'abord, nous considérons que la majorité électorale doit être fixée à un âge où l'expérience de la société et l'exercice de responsabilités doivent être avérés et témoigner d'une certaine maturité. L'âge de 16 ans ne permettrait pas toujours ce recul. Car voter, c'est assumer une part de responsabilités dans des choix collectifs qui engagent l'avenir de la collectivité. Tous les adolescents sont-ils en capacité de porter cette charge ? Ce n'est pas si sûr. Certains font valoir le fait que de nombreux droits sont déjà ouverts à l'âge de 16 ans ; néanmoins, nous ne pensons pas que participer à la création d'une association ni même voter aux élections prud'homales- pour les jeunes qui travaillent -est comparable avec l'expression du suffrage politique. De surcroît, on ne peut ignorer les raisons juridiques majeures qui s'opposent à l'abaissement de la majorité électorale prévu par l'article 1. Je rappelle que, conformément à l'alinéa 4 de l'article 3 de la Constitution, « sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». Ainsi, il est clair que la majorité électorale découle de la majorité civile et que les deux majorités ne peuvent être dissociées. vous n'ignorez pas qu'en 1974, lors de l'examen de son projet de loi, le gouvernement d'alors s'était appuyé sur l'avis du Conseil d'État pour considérer que la Constitution permettait d'abaisser l'âge de la majorité électorale indépendamment de celui de la majorité civile.

En outre, il était entendu à l'époque que le gouvernement souhaitait procéder par étapes, en commençant par abaisser l'âge de la majorité électorale, avant d'abaisser également l'âge de la majorité civile. Par conséquent, si nous souhaitions aujourd'hui abaisser l'âge de la majorité électorale, l'alternative serait la suivante : ou bien l'on révise la Constitution, ou bien l'on abaisse, de façon concomitante, l'âge de la majorité civile. de la majorité civile à 16 ans ne peut constituer une option, au regard des risques importants que cela comporterait pour la protection juridique et sociale des jeunes âgés de 16 à 17 ans

qu'une modification aussi substantielle du corps électoral ne saurait intervenir à quelques mois seulement du premier tour du scrutin présidentiel. En prévoyant une entrée en vigueur au 1 janvier 2022, l'article 5 de la proposition de loi serait ainsi contraire au principe de stabilité du droit électoral, que le Sénat a consacré il y a deux ans. Au demeurant, si nous étions prêts à consentir à une telle dérogation à ce principe, il serait impossible, de l'aveu même du ministère de l'intérieur, de procéder au recensement puis à l'inscription sur les listes électorales de 1,7 million de jeunes en l'espace de quelques mois. Enfin, au regard des études disponibles et des auditions menées, l'ouverture du droit de vote à 16 ans ne nous semble pas pertinente. Au contraire, d'après les enquêtes de l'IFOP, par exemple, une large part des jeunes estime aujourd'hui que la politique ne peut rien pour eux. C'est regrettable. Bien plus, pour beaucoup, l'exercice de la citoyenneté passe davantage par la participation aux manifestations et la signature de pétitions plutôt que par le recours aux outils traditionnels de la démocratie représentative. Du reste, il n'est pas tout à fait certain que l'ouverture du droit de vote aux jeunes âgés de 16 et 17 ans permette d'améliorer la participation des jeunes à moyen terme. Si la thèse selon laquelle les électeurs participeraient d'autant plus aux scrutins tout au long de leur vie qu'ils auraient commencé à voter jeunes est défendue par certains sociologues, elle est loin de faire l'unanimité. D'ailleurs, les précédents étrangers ne permettent pas de conclure au caractère incitatif de cette mesure. Ainsi, en Autriche, qui est l'un des trois seuls pays de l'Union européenne à avoir abaissé la majorité électorale en 2007 en deçà de 18 ans, cet abaissement n'a pas eu d'incidence notable sur la participation des jeunes âgés de 18 à 30 ans, alors même qu'une partie de ces jeunes avait voté à 16 ans en ayant bénéficié d'une préparation au vote depuis 2008. Ainsi, à l'heure actuelle, rien ne permet de penser que les jeunes de 16 et 17 ans iront davantage voter que leurs aînés de 18 à 24 ans et que, de surcroît, ils conserveront cette habitude tout au long de leur vie de citoyen. Dans ces conditions, il me semble que la priorité est d'inciter les jeunes déjà dotés du droit de vote à en faire usage. Nous sommes en effet

qui permet de diffuser les valeurs républicaines à l'école. Ainsi, dans le cadre scolaire, il apparaît préférable de s'appuyer sur les enseignements existants afin de former les citoyens de demain plutôt que de créer un nouvel enseignement obligatoire, comme le prévoit l'article 2 de la proposition de loi. L'enseignement en sciences politiques et en histoire de la vie française et européenne, que prévoit le texte, recouvre en effet largement les objectifs et le contenu de disciplines déjà enseignées du primaire au lycée, telles que l'histoire-géographie, mais aussi et surtout l'enseignement moral et civique. Ces deux matières sont

continu intégré au baccalauréat, ce qui me semble plus abouti que le dispositif proposé. Ainsi, les programmes actuels permettent d'ores et déjà de former les élèves au fonctionnement des institutions et aux enjeux de la démocratie. Par ailleurs, au sein de la société, il existe de nombreuses formes de participation civique destinées

nous est proposé, à titre principal, de rendre obligatoire la création d'un conseil de jeunes dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants et les départements. Je tiens à rappeler que les collectivités locales se sont déjà largement approprié ces dispositifs favorisant l'engagement citoyen des jeunes puisque près de trois quarts des régions et deux tiers des départements ont déjà institué de tels conseils. J'ai pu constater, comme vous, mes chers collègues, que de nombreuses communes, notamment depuis le dernier renouvellement des équipes municipales, s'engagent dans une telle démarche.

ce débat autour de la jeunesse parce qu'aucune question concernant la démocratie ou la jeunesse n'est anodine, encore moins ce qui touche à la citoyenneté. Il nous faut l'aborder avec rigueur parce que l'histoire de la démocratie est une histoire de conquêtes, de juste équilibre entre droits et devoirs, entre progressisme et conservatisme. Il est facile de balayer cette question en disant : « Oui, je suis pour ! » ou « Non, je suis contre ! », sans aller plus loin. loin. Ce serait bien méconnaître la question elle-même : dire oui ou non au vote à 16 ans, ce n'est pas dire oui ou non à la jeunesse, ce n'est pas donner les clés de la vie politique et institutionnelle à des adolescents et à des jeunes qui sont, pour les uns, force créatrice de notre pays, et, pour d'autres, encore des enfants n'étant pas en capacité d'exercer une responsabilité citoyenne. Ce n'est pas non plus résoudre d'un coup de baguette magique le problème endémique dont nous souffrons, et qui s'aggrave de plus en plus : celui de l'abstention.

Voilà pourquoi ils marchent pour le climat, signent des pétitions plus volontiers qu'ils ne votent. Toutefois, la démocratie, ce sont des droits mais aussi des devoirs. Et manifester sans voter revient à réclamer des droits sans s'imposer le devoir de les exercer et de décider.

Notre responsabilité est de former et d'accompagner les jeunes pour qu'ils connaissent le pouvoir du bulletin de vote, le pouvoir de la démocratie représentative, et qu'ils sachent exercer ce magnifique devoir démocratique. Former, comme nous le faisons, c'est renforcer l'éducation civique et morale, développer la démocratie scolaire, accompagner en construisant des parcours de citoyenneté. Car, oui, celle-ci s'apprend dès le plus jeune âge, elle s'apprend dans une expérience encadrée dans le temps scolaire ou extrascolaire. C'est l'expérience d'un jeune qui s'engage à l'école en tant que délégué de classe, en tant qu'éco-délégué, dans un conseil de la vie collégienne ou dans un conseil de la vie lycéenne. C'est l'expérience d'un engagement bénévole au travers d'une mission d'intérêt général, dans le cadre du service national universel (SNU), du volontariat, du service civique ou du corps européen de solidarité. C'est l'affaire des familles, c'est l'affaire de l'État et celle, également, de l'éducation nationale et des associations, mais c'est notre devoir de responsables politiques et d'élus. Je pense en particulier aux maires, qui sont en réalité ce lien le plus proche.

là où l'on comprend aisément que pour se soigner il faut des soignants et des hôpitaux, que pour se déplacer il faut des transports en commun, que pour se cultiver il faut des médiathèques, des salles de spectacle, et que tout cela dépend de nos choix.

autant que possible, à organiser des moments qui sacralisent ce rituel : des cérémonies citoyennes qui sacralisent la remise de la première carte électorale et qui matérialisent l'entrée effective dans la citoyenneté. Ces moments de vie, ces temps forts, ces temps forts, sont incontournables. Mesdames, messieurs les sénateurs, il ne vous aura pas échappé que, pour le moment, je n'ai pas définitivement répondu à la question. Mais je vais le faire. Ah ! Les conditions ne semblent pas réunies pour soutenir cette proposition d'abaisser l'âge de vote à 16 ans. Les enjeux, aujourd'hui, consistent à lutter contre l'abstention

cela peut paraître évident, mais ce ne l'est pas -, l'âge où le parcours d'apprentissage de la citoyenneté, dont la construction nous incombe, permet aux jeunes de revendiquer des droits mais aussi d'exercer les devoirs qui sont les leurs. Creuset républicain, mais aussi rite de passage, le service national universel est appelé à devenir un dispositif majeur de ce parcours d'apprentissage à la citoyenneté. Je suis convaincue que ce sera un accélérateur d'entrée dans la vie citoyenne active.

oubliant ainsi que l'avenir- notre avenir -est entre leurs mains. Je vous épargnerai le rappel de tout ce qui leur a été infligé ces dernières années, en particulier pendant la crise sanitaire sanitaire qui perdure. Ils avancent dans la vie dans un environnement incertain. Comment les mettre en confiance, alors que la politique s'écarte de son objet initial ? Comment les intégrer dans la vie de la cité ?

À mes côtés, de part et d'autre de la foule, les jeunes scandent des slogans très souvent accusateurs contre le système politique et, de fait, contre les personnes qui le composent. devons nous remettre en question en permanence ; nous devons nous ouvrir à cette jeunesse, qui ne demande qu'à être écoutée. Si le taux d'abstention record des 18-25 ans aux dernières élections est préoccupant, il convient d'interroger les raisons de ce désintéressement et de cette défiance.

On peut dès lors aisément concevoir qu'ils aient la capacité d'exprimer un suffrage éclairé. Il faut leur faire confiance. Abaisser le droit de vote à 16 ans, c'est permettre à cette jeunesse de s'investir pleinement et plus tôt. Donner les moyens d'un apprentissage solide en sciences politiques et en éducation civique constitue, j'en suis certaine, un très bon remède contre l'abstention. Je voterai pour ce texte.

la participation électorale s'effrite depuis 1989, les années 2020 et 2021 ayant constitué des records. Les jeunes figurent effectivement parmi les plus abstentionnistes, en concurrence avec leurs aînés de plus de 80 ans. Cette évolution est inquiétante : le vote, c'est la pacification de la vie politique ; l'alternative, c'est la participation violente. Dans ces conditions, il faut essayer de nouvelles solutions.

Deuxième argument : le risque d'effet domino sur d'autres majorités, qui viendrait diminuer la protection des mineurs. Il existe d'ores et déjà une pluralité de majorités et cette pluralité peut tout à fait être maintenue.

Le niveau d'éducation et d'accès à l'information des jeunes de 16 ans d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui des jeunes de 18 ans de 1974. Par ailleurs, un jeune sur cinq âgés de 16 à 18 ans a déjà participé, par exemple, à une marche pour le climat. Cette jeunesse aspire à des responsabilités et elle sait les prendre.

Aujourd'hui, à 16 ans, on peut payer des impôts, travailler, avoir des responsabilités associatives, exercer une autorité parentale, être poursuivi en justice. Vouloir disposer des mêmes droits démocratiques que les adultes semble cohérent. Une démocratie forte prend de meilleures décisions quand elle englobe l'ensemble du corps électoral et tient compte de la voix du plus grand nombre. Il est évident que le droit de vote à 16 ans permettrait à la jeunesse de donner son avis sur des thèmes qui la concernent au premier chef. D'objets politiques, les jeunes deviendraient des acteurs politiques. Bien entendu, la contribution de l'école, en tant qu'espace de socialisation politique, est essentielle, tout autant que la délibération dans des instances locales. C'est le sens des expériences conduites en Norvège et en Finlande. Jean-Pierre Raffarin relevait la permanence d'une méfiance de la part de vote envers ceux qui en sont dépourvus. Nous ne partageons pas cette méfiance. La jeunesse doit être prise au sérieux. Elle est digne de confiance. Sa voix compte. Elle peut et doit pouvoir prendre pleinement part à la conversation démocratique de notre pays. La

être en âge de porter plainte seul, de commencer à conduire, de faire un service civique ou de signer un contrat d'apprentissage ne signifie pas être en âge de voter. La citoyenneté se forme avec le temps, avec les expériences, les espoirs, la somme des ambitions et des échecs. L'enjeu va au-delà d'une nationalité, à laquelle on ajouterait une éducation et une somme d'années. Pourtant, en tant que législateurs, il nous faut bien fixer une limite, une frontière, un âge précis. Il existe, en fait, plusieurs majorités- électorale, civile, pénale -, qui sont aujourd'hui alignées. La majorité implique ainsi, à terme, une série de responsabilités particulièrement lourdes, mais aussi de devoirs, qui peuvent être autant de contraintes pour un jeune de 16 ans responsabilité judiciaire accrue, probité, possibilité de poursuites pour endettement ... La liste pourrait être longue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la proposition de loi propose de n'abaisser que la seule majorité électorale. électorale. L'abaissement du droit de vote à 16 ans n'est pas une demande émanant d'une majorité de mineurs. Elle procède plutôt d'une volonté politique, dans les nombreux termes d'un débat qui est d'ores et déjà posé. Une résolution du Parlement européen du 11 novembre 2015 « recommande aux États membres, pour l'avenir, d'envisager d'harmoniser l'âge minimal des électeurs à 16 ans, afin de garantir une plus grande égalité aux citoyens de l'Union lors des élections Plusieurs États européens fixent déjà le droit de vote à 16 ans : l'Autriche et Malte à l'échelle nationale, l'Écosse et une partie de l'Allemagne à l'échelle locale, la Slovénie sous condition d'emploi. On peut regretter, par exemple, que les jeunes qui sont particulièrement engagés, parfois adjoints et même maires, ne puissent pas se présenter en qualité de candidats à une élection sénatoriale pour laquelle ils sont, malgré tout, grands électeurs. La décorrélation entre l'âge de candidature et l'âge de vote est un autre sujet, dont notre chambre a souvent débattu. Aujourd'hui, gardons en tête qu'il s'agit de protéger nos jeunes. jeunes. Tous ne sont pas aussi engagés, aussi enthousiastes pour la chose publique, aussi documentés que ceux auxquels nous pensons tous, dans nos départements. de loi vise donc à abaisser de 18 à 16 ans la majorité électorale seule, dans le but de favoriser la participation. Elle ne néglige pas l'aspect éducatif, en proposant aussi d'introduire un enseignement obligatoire aux sciences politiques dès le collège.

Enfin, la stabilité du droit électoral, inscrite dans le code électoral sur l'initiative de notre collègue Alain Richard, et qui implique que le droit électoral ne soit pas modifié dans l'année qui précède le scrutin, Le texte soulève, certes, plusieurs questions importantes, notamment celle de l'abstention des jeunes. Lors de l'élection présidentielle de 2017, 21,3 % des personnes âgées de 18 à 24 ans inscrites sur les listes électorales n'ont voté à aucun des deux tours, contre 14,6 % de l'ensemble des électeurs inscrits. Aux dernières élections régionales, près de 87 % des 18-24 ans se sont abstenus au premier tour. Le phénomène d'abstention est réel. On peut douter de la faculté de cette proposition de loi à raviver mécaniquement la mobilisation de cette classe d'âge dans les urnes, laquelle reste pourtant le défi de fond qui se pose aux responsables politiques. C'est d'ailleurs dans le sens d'une réflexion approfondie et englobante que le Premier ministre a saisi le CESE, en septembre 2021, sur la participation des jeunes à la vie démocratique.

En 2022, plus de 200 000 jeunes pourront par ailleurs s'engager dans une mission de service civique. La lutte contre l'abstention est essentielle. À ce titre, l'inscription sur les listes électorales a été utilement facilitée pour lutter contre la mal-inscription.

au travers ce texte renforcer l'implication des jeunes dans la vie politique de notre pays, ainsi que Mme la rapporteure Nadine Bellurot pour son travail : tout en saluant le projet porté par nos collègues socialistes, elle a su préserver les équilibres nécessaires entre exigence constitutionnelle et liberté des collectivités territoriales.

de pré-majorité en vertu duquel les jeunes âgés de 16 et 17 ans seraient autorisés à voter aux élections municipales. À l'Assemblée nationale, pas moins de trois propositions de loi ont visé à ouvrir le droit de vote aux jeunes de 16 ans pour toutes les élections. cela a été rappelé, des recommandations ont également été émises en ce sens par le Parlement européen. Chaque fois, les idées n'ont pas été suivies d'actes. L'abaissement de la majorité électorale à 16 ans tel que prévu à l'article 1 de cette proposition de loi concernerait près de 1,7 million de nos jeunes concitoyens et entraînerait une augmentation de l'effectif du corps électoral de près de 3,5 %. Cette augmentation serait importante, certes, mais dans les faits peu efficace. Aujourd'hui, notre jeunesse se sent désintéressée par le vote, non par la politique. Elle exprime ses revendications par le recours à d'autres modes d'expression, comme les manifestations, les pétitions ou des initiatives ciblées. Avant de faire voter les moins de 18 ans, nous pourrions commencer par tenter de ramener aux urnes ceux qui détiennent aujourd'hui le droit de vote. Abaisser le droit de vote à 16 ans supposerait une révision de la Constitution. Comme l'a indiqué justement notre rapporteure, l'alinéa 4 de son article 3 dispose que « sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». Autrement dit,

Ces impossibilités, tant pratiques que constitutionnelles démontrent qu'accorder le droit de vote dès l'âge de 16 ans n'est, aujourd'hui, pas réalisable. L'autre mesure de cette proposition de loi doterait les communes de plus de 5 000 habitants d'un conseil de jeunes.

La création d'une nouvelle instance remettrait en question la nécessaire liberté dont les collectivités territoriales disposent pour favoriser la participation des jeunes aux décisions locales. La commission des lois, bien qu'ayant rejeté l'ensemble du texte, juge cependant préférable de s'appuyer sur l'existant pour renforcer l'engagement des jeunes et les accompagner dans l'exercice de leur citoyenneté. Les auteurs de la proposition de loi entendaient introduire un enseignement obligatoire aux sciences politiques et à l'histoire de la vie française et européenne dès l'entrée au collège. Aujourd'hui, l'enseignement moral et civique, l'histoire-géographie et les sciences économiques et sociales- matières déjà présentes dans le corpus scolaire - peuvent répondre à cet objectif, en formant les élèves au fonctionnement des institutions. Les programmes scolaires

d'accompagner ces jeunes dans l'apprentissage de la citoyenneté en amont et, en parallèle de leur accession à la majorité, de leur proposer d'autres formes d'engagement, notamment associatives, possibles à tout âge, ou encore la possibilité d'effectuer un service civique.

qui estime, à juste titre, que « la collectivité publique doit [ ...] privilégier vis-à-vis des futurs citoyens un accompagnement leur permettant de mesurer, à leur majorité, la responsabilité qui leur incombe dans la participation aux choix politiques ». C'est pourquoi

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, dont je salue le « baptême du banc », mes chers collègues, personne ici n'ignore la crise démocratique, cette fonte des glaces citoyennes qui fragilise nos institutions, affaiblit la légitimité des élus et exprime une perte de confiance durable envers les responsables politiques et la parole publique. Chez les jeunes, cette défiance semble structurelle. Chaque rendez-vous électoral en donne la triste démonstration, si l'on en juge par les taux d'abstention record bien plus élevés que chez leurs aînés. Ce constat, nous l'avons en partage avec les auteurs de cette proposition de loi. Pourtant, le texte que nous examinons offre-t-il un remède à la hauteur du péril du désenchantement démocratique français ? J'en doute fort. Comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, cette proposition de loi est porteuse de néfastes confusions. Il suffit de lire le premier paragraphe de l'exposé des motifs pour découvrir sa logique pour le moins audacieuse. Puisque les jeunes votent moins, faisons-les voter plus tôt, dès 16 ans Comprenne qui pourra la subtilité de cet étrange syllogisme ! On connaissait le pari de Pascal, on découvre celui des sénateurs socialistes. Loin de se restreindre à une simple réforme des dispositifs existants, ce texte bouscule le concept de citoyenneté lui-même. Car que Car que signifierait la fin de l'ouverture du droit de vote à l'âge de la majorité civile ? Que donnerait-elle à voir ? Le droit de vote étant inséparable de la majorité civile, 1,5 million d'adolescents seraient invités à se rendre aux urnes, alors même qu'ils sont reconnus comme largement irresponsables par le droit français. Ces jeunes jouiraient alors d'un droit politique majeur, sans être astreints à l'ensemble des devoirs impliqués par la citoyenneté. Cherchez l'aberration ! Mes chers collègues, en souhaitant abaisser le droit de vote à 16 ans, vous vous référez à certains droits acquis à cet âge, comme la conduite accompagnée ou l'accès C'est oublier que l'accès au vote renvoie à la citoyenneté et qu'il suppose une responsabilité d'une tout autre nature. Victor Hugo évoquait, lors d'un discours formulé en mai 1850 sur le suffrage universel, ce ce droit de suffrage qui « fait partie de l'entité du citoyen, ce droit de suffrage sans lequel le citoyen n'est pas ». Ce lien essentiel, votre texte entend aujourd'hui le briser, séparant le plus fondamental des droits politiques de la plus belle des qualités, celle de citoyen français. Pis, vous dissociez le droit de vote de celui d'éligibilité. On pourrait donc élire à 16 ans, mais n'être pas soi-même éligible. Vous créeriez ainsi des « pré-citoyens » ou des citoyens hybrides. À cet égard, on jugera d'autant moins opportun de voter une mesure d'une telle portée dans le cadre d'une simple niche parlementaire, sans même songer à l'inévitable problématique constitutionnelle qu'impliqueraient les dispositions qu'elle contient. Quant aux programmes scolaires en résonance avec le fait citoyen, il en va comme de la loi, selon la célèbre formule de Montesquieu : « Il n'y faut toucher que d'une main tremblante.

Pourquoi alourdir artificiellement le bréviaire de nos professeurs, alors même que les élèves sont d'ores et déjà invités à penser les formes d'engagement politique, social et associatif ? Permettez-moi également de douter des sciences politiques que l'on prétend, par ce texte, introduire au collège, discipline dont l'objectivité pourrait être dévoyée par l'idéologie. L'école, le collège, le lycée doivent contribuer à éveiller, à former la conscience de futurs citoyens éclairés, pas à embrigader de futurs militants espérés. Ce n'est pas seulement, comme cette proposition de loi le postule, parce qu'un adolescent de 16 ans est antiraciste, féministe ou animaliste qu'il doit pouvoir exercer le droit de vote. Enfin, pour mieux enraciner la citoyenneté dans notre jeunesse, votre texte prévoit la création obligatoire d'un conseil municipal de jeunes dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants et dans les départements. Oui aux conseils municipaux de jeunes, qui peuvent se révéler être de remarquables centres de formation d'apprentis citoyens, tout en faisant jaillir quelques salves d'idées rafraîchissantes, mais certainement pas de façon imposée l'obligation dénature, dévalorise et décourage toujours l'intention. Quand un droit devient un devoir, la magie se mue en mécanique. On fait parce qu'il faut faire, non parce qu'on a envie de faire.

La liberté n'est-elle pas le pilier de notre pacte républicain ? Avez-vous oublié les libertés des collectivités locales ? Arrêtez de vouloir les caporaliser et de forger de nouveaux carcans ! Faites confiance à l'imagination, à la volonté d'écoute et à la capacité d'innovation des élus locaux. Ils n'ont pas besoin du législateur pour avoir à coeur d'impliquer la jeunesse de leur territoire. Ils mesurent, comme nous, la valeur de cet engagement. Dieu merci, le texte ne prévoit pas d'éventuelles amendes pour les municipalités rebelles à ce possible diktat Il n'en restera pas moins vain, pour ne pas dire contre-productif. Aux antipodes de cette proposition ubuesque, un dispositif comme le service civique- vous y êtes attachés, -permet aujourd'hui, dès l'âge de 16 ans, de s'investir au service de l'intérêt général et d'engager une approche ô combien formatrice des valeurs et principes inhérents à la citoyenneté. C'est précisément ce type de dispositif qui mériterait d'être poursuivi, amélioré et, pourquoi pas, développé. En définitive, même si les intentions de ses auteurs se voulaient vertueuses, cette proposition de loi se révèle être bien pauvre et décevante. Elle n'est, en fait, qu'un médiocre exercice d'affichage politique du parti socialiste à l'endroit d'un électorat convoité. Loin de comporter un véritable remède au désengagement, elle n'offre pas davantage matière à revitaliser la culture civique de notre jeunesse. C'est dans cet esprit que le groupe Les Républicains s'y opposera. Quelle surprise

Vogel. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, notre pays vieillit- c'est une réalité démographique -et la jeunesse est de plus en plus angoissée par la crise climatique et sociale qui assombrit son avenir.

82 % des moins de 35 ans se sont abstenus lors des dernières élections régionales, contre 66,7 % pour l'ensemble des électeurs. Il s'agit là de deux records absolus sous la V République. Pourquoi ce paradoxe ? Pourquoi une génération si inquiète pour son avenir ne prend-elle pas davantage part au choix des responsables qui en décideront ? La jeunesse qui ne vote pas serait-elle, comme on l'entend souvent, dépolitisée, désabusée, irresponsable ou démobilisée ? Rien n'est moins faux. La jeunesse de notre pays est plus politisée que jamais : elle manifeste pour le climat, contre les violences policières ; elle s'investit dans des associations féministes, de protection de l'environnement, pour le bien-être animal ; elle invente de nouvelles façons de consommer qui sont plus éthiques, plus responsables.

tant que les priorités des gens seront le pouvoir d'achat et la planète, tant que l'on discutera de laisser ou non mourir des migrants, ou du menu des réceptions officielles de la ville de Grenoble, ils n'auront pas l'impression qu'il est utile de s'impliquer ! Il faut donc impérativement recentrer le débat public sur les vrais problèmes du siècle : la crise climatique, les nouvelles solidarités, la refondation démocratique.

Mais c'est aussi la décision politique elle-même qu'il faut changer. Il faut que nous, politiques, partagions notre pouvoir avec les citoyens. Des modes de démocratie plus directe, plus locale, plus participative, plus collaborative,

des horizons indépassables, les seuls indicateurs de la participation citoyenne. Cela étant dit, le sujet qui nous occupe aujourd'hui est plus restreint : il s'agit simplement d'ouvrir le droit de vote à 16 ans. de vous expliquer pourquoi les écologistes y sont favorables. Personne n'a dit que cette solution était la seule et l'unique, ni qu'à elle seule elle résoudrait tout. Mais elle va dans le sens de l'Histoire. Il faut que la jeunesse nous demande des comptes,

Par ailleurs, les travaux de sociologie le montrent : plus les jeunes attendent pour participer à la vie politique, moins ils s'engagent à l'âge adulte. Voilà pourquoi nous n'avons plus le temps d'adresser une fin de non-recevoir aux demandes d'implication politique de la jeunesse. Le groupe écologiste votera

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, « comme un baromètre, le niveau d'abstention est un indicateur du climat de l'opinion, du lien entre les citoyens et leur représentation politique, et plus largement de l'état de santé du système démocratique ». Ces mots de la sociologue Anne Muxel, spécialiste de la participation politique, datent de 2007- ils résonnent d'autant plus aujourd'hui. Nous constatons à chaque élection un taux d'abstention particulièrement fort et les jeunes sont parmi les premiers à ne pas se diriger vers les urnes. Si l'élection présidentielle mobilise toujours, toujours, la participation des 18-24 ans est inférieure en 2017 à la moyenne générale. Ce taux s'effondre à 31 % pour les élections législatives, puis à 28 % pour les élections municipales et enfin à 17 % pour les dernières élections régionales et départementales En tant que représentants de la République, ces chiffres ne peuvent que nous accabler et nous partageons l'objectif de cette proposition de loi de lutter contre l'abstention massive de nos jeunes. Mais la réponse de nos collègues du groupe SER correspond-elle à la bonne question, à ce problème que nous identifions toutes et tous ? Nous ne le pensons pas. Avant toute chose, nous tenons à dire que nous ne sommes pas opposés à encourager la participation politique des moins de 18 ans. Les dernières grandes manifestations pour le climat, les droits des femmes ou la lutte contre le racisme ont été de tels succès grâce à la présence de ces jeunes. Ce que nous ne partageons pas, c'est le raccourci entre le problème de l'abstention et l'élargissement de l'électorat à une population plus jeune, qui elle-même ne le demande pas. Pire, une telle proposition entretient la confusion entre les droits et devoirs rattachés à la majorité électorale et ceux rattachés à la majorité civile et pénale. ces majorités risquerait d'affaiblir la protection actuelle des mineurs, dont la responsabilité pénale est atténuée concernant les sanctions et pour lesquels peuvent être décidées des mesures d'assistance ou d'éducation. Nous ne sommes plus dans le même débat que dans les années 1970, où était en jeu un abaissement plus général de la majorité civile. L'abstention des jeunes nous renvoie à l'état de notre démocratie, à l'état du lien entre les citoyens et leurs représentants. Ce lien est aujourd'hui abîmé. Pour ramener les plus jeunes électeurs aux urnes, il faut susciter leur intérêt politique ; cela passe par les politiques publiques que nous votons et qui ne sont pas assez orientées vers ce public, ses besoins et ses attentes. Avant de se lancer sans crier gare dans un élargissement de l'électorat, attelons-nous à rapprocher la politique des électeurs actuels. Ces dernières années a été dénoncé le manque de transparence de la vie politique et de reconnaissance des électeurs ou du vote blanc. Le droit de vote ne fait pas tout, il ne s'entretient pas par le seul fait d'exister. La croyance en son utilité est essentielle, tout comme l'apprentissage de ce rituel républicain. Comme l'explique la sociologue Céline Braconnier, « si on se contente d'abaisser l'âge sans interroger le rôle de l'école, on risque de ne faire qu'augmenter l'abstention ». À ce titre, nous défendons le développement de lieux et de moments où l'éducation politique C'est par les libertés citoyennes et politiques que se forge l'opinion des jeunes, et nous sommes contre le musellement de l'expression des élèves dans les cours des lycées, élèves auxquels l'article L. 511-2 du code de l'éducation demande aujourd'hui une « neutralité » qui est bien illusoire. Nous ne pensons pas que les articles 2 et 3 de cette proposition de loi puissent apporter quelque chose de nouveau. Plutôt que d'alourdir de manière répétitive les programmes existants, il conviendrait de revaloriser l'enseignement moral et civique qui ne représente que trente minutes par semaine. Les objectifs cités dans ce texte sont déjà censés être largement couverts et la proposition qui nous est faite peut être vue comme une défiance envers le corps enseignant, lequel fait pourtant au mieux avec les moyens qui lui sont attribués et qui sont malheureusement si faibles. La normalisation de la participation électorale permettrait aussi de rendre l'acte de vote plus naturel. En France, les échéances électorales sont espacées et les citoyens sont finalement peu sollicités en comparaison, par exemple, avec le système suisse et ses référendums. La proximité des élections présidentielle et législatives a aussi fait perdre de la valeur à ces dernières élections, souvent considérées comme une simple validation de la première. Enfin, je voudrais évoquer le phénomène de la mal-inscription ou de la non-inscription sur les listes électorales, qui a concerné 13 millions de personnes en 2017. Ce sont les citoyens les plus mobiles qui sont particulièrement concernés, ainsi que les étudiants et les jeunes. Ne pas être inscrit dans le bureau de vote de sa commune multiplierait par trois le risque d'être un abstentionniste constant. La réforme de l'inscription va dans le bon sens, en permettant un allongement des délais, mais d'autres dispositifs sont à trouver pour faire du vote non pas un fardeau administratif, mais bien un droit des citoyens inhérent à leur quotidien. Pour toutes ces raisons, nous voyons en cette proposition de loi un appel à lutter contre l'abstention, mais la solution de nos collègues manque son objectif. C'est pourquoi le groupe CRCE ne votera pas ce texte. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'abstention suscite des craintes bien légitimes, car chaque fois qu'elle progresse, c'est la démocratie qui s'affaiblit et qui recule. Malheureusement, depuis plusieurs décennies, notre vie électorale est marquée par une abstention récurrente. Si dans les années 1970, la participation était supérieure à 80 %, l'abstention a depuis progressé de façon régulière pour dépasser aujourd'hui Seule l'élection présidentielle semble échapper, pour le moment, à cette tendance. Elle reste l'élection qui enregistre les taux de participation les plus élevés. Néanmoins, au premier tour du scrutin présidentiel de 2017, un tiers des 18-25 ans n'a pas voté. Plus récemment, lors des élections départementales et régionales de juin 2021, plus de 60 % des électeurs ne se sont pas déplacés et ces chiffres ont atteint 86 % chez les jeunes. Devant ce constat d'affaiblissement de la participation électorale, de nombreuses initiatives parlementaires ont vu le jour. vu le jour. Ainsi, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi entend apporter une solution à l'abstention massive des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Elle vise notamment à ouvrir le droit de vote dès l'âge de 16 ans et à instituer des conseils de jeunes dans les communes de plus de 5 000 habitants, ainsi qu'au sein des conseils départementaux. Les dispositions de ce texte appellent plusieurs remarques. Tout d'abord, la majorité électorale et la majorité civile sont fixées à 18 ans depuis la loi du 5 juillet 1974 et l'ouverture du droit de vote à 16 ans

Enfin, les dispositions visant à renforcer les obligations pesant sur les collectivités territoriales en matière de conseils de jeunes sont, à mon sens, malvenues. Bien au contraire, il apparaît primordial de sauvegarder l'initiative et l'autonomie des élus municipaux et départementaux en la matière. L'article 55 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté prévoit d'ores et déjà qu'une collectivité territoriale ou un EPCI peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de la jeunesse. Faisons confiance aux élus pour faire participer les jeunes de leur territoire à la vie démocratique, sans les étouffer par des contraintes excessives.

défiance vis-à-vis de la classe politique, mise en cause de la démocratie représentative, perte de confiance à l'égard des institutions, multiplication des inquiétudes quant à l'avenir, qu'il s'agisse de la crise sanitaire, du réchauffement climatique ou encore des nombreuses fractures qui fragilisent nos sociétés, les explications sont multiples et le diagnostic est aujourd'hui bien établi pour éclairer la crise citoyenne qui affecte notre pays et touche davantage encore les plus jeunes de nos concitoyens. Je suis de ceux qui pensent que toute initiative qui poursuit l'objectif de trouver des remèdes à cette crise mérite d'être soulignée et encouragée. Pour répondre à notre collègue Arnaud de Belenet, j'ai moi-même déposé en janvier dernier une proposition de loi pour rendre le vote obligatoire,

J'en suis persuadé, c'est par la conjonction de nos propositions, la confrontation de nos idées et la convergence de notre volonté commune de recréer cette conscience politique et citoyenne, qui fait cruellement défaut et met en danger notre République, que nous parviendrons à infléchir cette courbe préoccupante, pour ne pas dire dangereuse. oui, j'entends les objections de notre rapporteure sur les risques attachés à la décorrélation entre la majorité civile et la majorité civique et sur la nécessité d'en passer par une révision constitutionnelle. Oui, je comprends ses réserves quant à la préservation de la liberté des collectivités et à la nécessité de leur faire confiance pour renforcer l'implication des plus jeunes dans leurs instances participatives. Et oui, les programmes scolaires prévoient déjà l'enseignement des bases de notre système politique et de l'histoire de nos institutions. Mais force est de constater que ce n'est pas suffisant. Tant s'en faut ! Les causes de cette crise sont multiples et les solutions doivent l'être aussi. Pour utiliser une expression devenue commune aujourd'hui, ne faut-il pas provoquer un choc de la citoyenneté ? N'est-il pas temps d'en passer par plus d'encadrement, voire de contraintes, pour accompagner cette transformation nécessaire de notre société ? Sauf à considérer que ce déclin du fait politique n'est pas réversible, ce à quoi je ne me résigne pas ! Je sais parfaitement que la citoyenneté ne se dicte pas et qu'elle doit se construire par un travail de conviction et d'explication, par une compréhension de ses enjeux, par une conscientisation des combats et des sacrifices qui ont permis à chacun de pouvoir aujourd'hui exercer ses droits de citoyen libre et éclairé. Mais chacun sait aussi les dangers qui guettent notre démocratie. Une échéance électorale fondamentale se profile et nous voyons tous se multiplier les discours extrêmes, les provocations et les incitations à accroître les fractures et les tensions. La crise démocratique devient pour certains un argument de campagne et alimente le climat nauséabond de « dégagisme » général, porté par ceux qui se disent en dehors du système, mais dont le seul but est de le conquérir Il est de notre responsabilité de montrer à nos concitoyens que les élus de la République ont pleinement conscience de ces problématiques et qu'ils s'en emparent pour tenter d'y apporter des réponses, aussi imparfaites et insuffisantes soient-elles

à 16 ans, la maturité et l'autonomie sont déjà très avancées et c'est un âge auquel des responsabilités importantes sont déjà attachées- possibilité de travailler, apprentissage de la conduite, responsabilité pénale, engagement bénévole, etc. D'autres pays se sont déjà engagés sur cette voie et le Conseil de l'Europe s'y déclare favorable.

J'étais interpellé mercredi dernier par les mots que vous avez prononcés ici même. Je vous ai écouté vous enorgueillir de votre bilan à l'égard de la jeunesse : à vous entendre, vous auriez tout fait et tout bien fait. Oui, la jeunesse est insaisissable. Elle est diverse. Cependant, les faits sont têtus. Avant même la crise du covid, le Secours catholique relevait que le niveau de vie des 15-34 ans s'était très largement dégradé au regard du seuil de pauvreté. N'avez-vous pas vu ces milliers de jeunes faire la queue à la soupe populaire ? Que répondez-vous ? Vous baissez les aides personnalisées au logement et vous leur refusez un revenu minimum que nous avons proposé. Nombre d'études montrent aussi que la jeunesse perd le paradigme du collectif, c'est-à-dire de l'État, des partis politiques, des syndicats, qui n'appartiennent pas à leur mémoire collective. Vous faites mine de vous en étonner. Cette jeunesse partage pourtant un engagement commun : la protection de la planète. Qu'avez-vous fait ? Une loi Climat bien en deçà de ce que réclame la cause, un simulacre de participation citoyenne et pas une place accordée aux jeunes dans le débat. Les jeunes ne sont plus que 11 % à considérer qu'ils peuvent avoir une influence réelle sur les destinées de la France, selon la dernière étude de Frédéric Dabi, intitulée. Entre Entre les jeunes qui occupent des postes moins qualifiés que leurs parents et des emplois disponibles inférieurs au niveau de formation, la désillusion est très grande. Que leur proposez-vous ? L'entrepreneuriat individuel, l'ubérisation, la précarisation ... Le Président de la République n'a-t-il pas dit lui-même que travailler pour Uber soixante ou soixante-dix heures en touchant le SMIC permettait au moins d'entrer dans la dignité ? Et vous, tranquillement, vous considérez qu'avec des demi-mesures comme les vacances apprenantes, la rénovation de quelques logements, un chèque psy, le BAFA ou un contrat d'engagement, assumé comme une pâle copie de la garantie jeunes, vous répondez aux aspirations de la jeunesse. Mais quelle société leur proposez-vous ? C'est le coeur du problème Selon l'Insee, les syndromes dépressifs chez les 18-29 ans sont en forte augmentation. Le niveau de bonheur s'effondre, selon Frédéric Dabi. En 2021, 42 % des jeunes de 18 à 30 ans déclarent nécessaire d'avoir un idéal pour vivre : ce chiffre n'a jamais été aussi bas il était deux fois plus élevé il y a seulement vingt ans. La chute est vertigineuse. La jeunesse partage majoritairement la conviction que le monde tel qu'il est va vers une forme inconnue de désastre. La société que vous leur proposez est un monde où les jeunes sont sommés de gagner une place dans la compétition planétaire, un monde qui oppose celles et ceux qui bénéficient du système à celles et ceux qui ne parviennent pas à y entrer. À l'arrivée, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien, comme l'explique le Président de la République qui exhorte les jeunes Français à vouloir devenir milliardaires en traversant la rue ... L'impératif de réussite s'est imposé. Performant, compétitif, flexible, souvent issu d'un milieu culturellement favorable, tel est le profil du jeune « » dans la perspective darwinienne de l'économie libérale que vous proposez et que vous revendiquez depuis le premier jour- je vous le reconnais. L'individu que vous voulez est non pas un coopérateur, mais un compétiteur. Ce système est une machine à broyer la solidarité, un système que vous appuyez sur l'illusion méritocratique : « quand on veut, on peut », tel est votre mantra. Vous considérez qu'au fond celui qui « réussit », c'est parce qu'il en a les qualités il s'est efforcé d'y parvenir et donc il a une dignité supplémentaire par rapport à celui qui n'a pas « réussi », parce qu'il serait paresseux, incompétent, sans talent. C'est une analyse erronée qui vous permet de dire aux individus qu'ils sont seuls responsables de leur destin, et de mettre en oeuvre des politiques conservatrices plutôt que de remettre en cause ce déterminisme social et

Le scrutin est ouvert.

Merci